Madame la présidente,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

Au cours de la discussion de l'article 9 relatif à la suppression de petites taxes, les députés ont souhaité procéder, par voie d'amendement, à la suppression de la taxe sur les friches commerciales.

des locaux vacants et à permettre d'engager un dialogue avec les propriétaires de ces locaux. Alors que les plans de revitalisation de centre-ville se multiplient sur le territoire, notamment sous l'impulsion du plan », qui a été initié par le Gouvernement et qui était porté par le ministre Jacques Mézard, il nous paraît particulièrement inopportun de supprimer ce levier fiscal. Nous proposons donc de revenir sur la mesure adoptée par l'Assemblée nationale.

La taxe dite « TA-IFER », prévue par l'article 1609 du code général des impôts, est une contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l'IFER, applicable aux stations radioélectriques- c'est donc une taxe sur les antennes de téléphonie portable. Le produit de cette taxe- 8,4 millions d'euros en 2018 -permet de financer les mesures des champs électromagnétiques émis par les stations, ainsi que la recherche sur leurs effets sur la santé humaine. La taxe vise à mettre en oeuvre les orientations retenues dans le cadre du Grenelle de l'environnement : l'article 42 de la loi du 3 août 2009 a en effet prévu la mise en place d'un dispositif de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques, conduit par des organismes indépendants accrédités. Ce dispositif doit être financé par un fonds indépendant alimenté par la contribution des opérateurs de réseau émettant des ondes électromagnétiques. L'objectif de simplification et de réduction de la pression fiscale visé par l'article

ont clairement mis en évidence la nécessité des contrôles et de la poursuite des recherches, en maintenant leur financement sous une forme indépendante et pérenne. Cet amendement vise à préserver le produit de cette taxe, qui contribue au budget de l'État à hauteur de 3,5 millions d'euros, à l'Agence est chargée du financement de la recherche sur les effets sur la santé des champs électromagnétiques, dans la limite de 2 millions d'euros, et à l'Agence nationale des fréquences, l'ANFR, qui est chargée du financement de la mesure des champs électromagnétiques, dans la limite de 2,9 millions d'euros.

Le projet de loi de finances prévoit la suppression de la taxe hydraulique affectée à Voies navigables de France, VNF, et son remplacement par un régime de redevances domaniales de droit commun. Le présent amendement vise à maintenir le mécanisme actuellement appliqué, qui permet aux titulaires d'ouvrages notamment d'assainissement et liés à la production d'eau, de répercuter tout ou partie du montant de la taxe hydraulique sur l'usager final du service, par l'application d'un supplément au prix du mètre cube d'eau.

Ce dispositif, qui répondait à une simplification et à une plus grande lisibilité de la fiscalité locale, s'est accompagné, d'une part, d'un élargissement de son assiette puisque tous les supports publicitaires sont visés, y compris les enseignes, d'autre part, d'une révision à la hausse de ses taux. Le produit de la TLPE est devenu très dynamique, passant de 28,1 millions d'euros en 2007 à près de 183 millions d'euros en 2018, soit une augmentation de 551 %. Cette taxe, qui ne s'applique pas à toutes les formes de distribution- je pense à l'e-commerce -nourrit également de nombreuses critiques sur l'équité et l'égalité devant l'impôt. Qui plus est, les différences entre les communes ont alimenté la défiance des entreprises concernées. En effet, bon nombre de PME déplorent que la TLPE, à l'origine facultative, puisse s'appliquer dans un objectif de rendement et, dans certains cas, sans information préalable. La suppression, à terme, de la taxe d'habitation, votée dans le cadre de la loi de finances pour 2018, ne fait que renforcer les craintes des chefs d'entreprise quant à un rehaussement de la TLPE puisque cette dernière est également perçue au seul profit des communes. C'est pourquoi, puisque le Gouvernement souhaite

réguler et de faire en sorte que le paysage urbain ne ressemble pas à tout et n'importe quoi. De plus, c'est un fait que cette taxe, qui en a remplacé d'autres, finalement, rapporte de l'argent. Ce n'est peut-être pas le moment de venir supprimer des ressources propres à nos communes.

1,1 % appliqué lors du partage d'un bien ou d'une licitation. Nous avions adopté l'an dernier la première partie de cet amendement,

n° I-603 rectifié. Cet amendement concerne les concessions de barrages hydroélectriques pour lesquelles, chacun le sait, les concessionnaires versent une redevance à l'État et aux collectivités locales.

au milieu du XX siècle. S'il fallait les construire aujourd'hui, je ne doute pas que de nombreuses associations nous expliqueraient qu'ils ne produisent pas une bonne énergie renouvelable. Il n'en demeure pas moins qu'ils constituent un atout pour la France. Nous avons fait depuis

Je ne peux pas laisser passer ce débat sans dire la gravité du choix fait pour l'avenir de rouvrir la concurrence sur les concessions. Je reste convaincue que l'énergie hydroélectrique doit demeurer dans le service public,

dans les objectifs ambitieux que la France doit poursuivre sur l'ensemble de son territoire au bénéfice des énergies renouvelables, dont l'énergie hydroélectrique, qui bénéficie de nombreux avantages et doit être promue. je ne fais pas la publicité de ce qu'a dit hier le Président de la République. Celles et ceux qui partagent une ambition écologique en faveur des énergies renouvelables doivent, à l'évidence, s'inscrire complètement dans cette démarche.

les étudiants en recherche d'emploi après avoir obtenu en France un diplôme de niveau master et les étudiants relevant d'un programme de mobilité européenne. Tous sont assujettis, dans le cadre des dispositions en vigueur du à une taxe fixée au tarif maximal pour la délivrance de leur titre de séjour. Ces publics ayant des revenus limités, il est proposé, dans une logique d'attractivité, de les assujettir à des tarifs minorés. Par comparaison, les étrangers titulaires d'un titre de séjour étudiant bénéficient déjà d'un tarif minoré.

Je fais le diagnostic d'une politique de Gribouille sur l'ensemble de ce dispositif

! Cet amendement vise à plafonner le montant des taxes que les étrangers doivent acquitter lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'un premier titre de séjour ou le renouvellement d'un titre de séjour. Ce montant maximal est aujourd'hui de 269 euros, soit une taxe de 250 euros pour l'octroi du titre et un droit de chancellerie de 19 euros.

Afin de pouvoir payer les sommes qui leur sont réclamées, de nombreux migrants sont contraints de demander de l'aide à leurs proches ou à des associations ; certains préfèrent même rester dans la clandestinité. nous proposons de fixer à 150 euros le montant maximal de la taxe relative à l'octroi d'un premier titre de séjour, de fixer à 87 euros celui de la taxe de renouvellement et de supprimer le droit de visa de régularisation.

taxe de chancellerie avait pour objectif principal de sanctionner financièrement les personnes qui n'avaient pas demandé un visa pour entrer en France alors qu'elles en avaient l'obligation, en leur faisant payer le double du prix du visa.

ou encore ayant pénétré légalement en France sous couvert d'un document délivré par un État membre de l'Union européenne se voient désormais exiger un paiement de 340 euros en sus des autres taxes liées au motif du séjour invoqué.

: La parole est à M. Xavier Iacovelli. Cet amendement a pour objet de supprimer le paiement d'une taxe de 50 euros, correspondant à une partie du droit de visa de régularisation, devant être effectué au moment même de la demande de titre de séjour, cette somme n'étant pas remboursable en cas de rejet de la demande. Cette disposition, introduite par la loi de finances pour 2012, constitue un véritable droit d'entrée dans la procédure d'admission au séjour. Elle n'a d'équivalent dans aucune autre procédure administrative effectuée en France. De ce fait, elle constitue une anomalie fiscale cantonnée au code de l'entrée et du séjour des étrangers

! On n'octroie pas de crédits suffisants à l'OFII pour l'intégration, pour le droit au logement, ou surtout pour faire en sorte que ceux qui obtiennent réellement le statut de réfugié

On ne peut pas ainsi amputer le budget de l'État à tout bout de champ et dans tous les domaines. Je regrette que vous n'ayez pas évalué le coût de cette mesure que vous proposez à notre vote. Pour le reste, naturellement, je suis fondamentalement opposé à ces amendements.

: elle permet de flécher des ressources sur des types de financement qui ne sont pas forcément très compatibles avec le principe de l'annualité budgétaire. Lorsqu'on finance une grande infrastructure, qu'elle soit ferroviaire ou routière,

à respecter des programmes d'infrastructure. En réalité, l'AFITF est l'enfant illégitime des amours contrariées du ministère de l'équipement et de Bercy. Le ministère de l'équipement obtient en général un peu d'argent pour des infrastructures, et Bercy le lui reprend.

et je lui demande de réactiver l'AFITF. Cette agence a l'immense mérite d'être un lieu où les dépenses d'infrastructure sont défendues, alors qu'elles servent en général de marge d'ajustement pour les gouvernements en difficulté. Rappelons-nous qu'il n'y a aucune raison que les gouvernements à venir ne soient pas, à leur tour, en difficulté

le problème de nos infrastructures. Chacun peut constater l'état de certaines routes ; il y a de moins en moins de routes nationales, et ce sont les collectivités territoriales qui doivent procéder aux travaux de renforcement et d'entretien. Quant

ce que Bruno Le Maire a annoncé le 27 avril 2011 : « Le Fonds d'aménagement numérique des territoires, FANT, a, quant à lui, été créé par la loi relative à la lutte contre la fracture numérique de décembre 2009. Il a pour objet de contribuer au financement de projets publics de déploiement du très haut débit conduits dans les zones qui ne font pas l'objet de déploiements privés. Il sera mis en oeuvre, une fois les crédits du programme des investissements d'avenir épuisés. Pour donner suite à cette affirmation, constatant, selon les propres dires des services de l'État et du Gouvernement, l'épuisement des crédits du Fonds national pour la société numérique, le FSN, il est proposé de créer une contribution de solidarité numérique, fixée à un euro par mois sur les abonnements à haut débit et à très haut débit et destinée à alimenter le FANT, qui permettrait d'achever les déploiements des réseaux en fibre optique pour 100 % de la population, des entreprises et des administrations françaises.

de solidarité sur les abonnements. Il s'agit là de créer une contribution de solidarité numérique sur les mobiles multifonctions haut et très haut de gamme. Alors que l'Europe cherche comment taxer les géants du net et qu'Apple est devenu spécialiste de l'optimisation fiscale, il ressort des études récentes que le prix d'achat moyen des smartphones augmente de façon sensible : la valeur globale du marché augmente elle

Plusieurs études ont d'ailleurs montré que, même si les ventes diminuaient, les prix d'achat continuaient d'augmenter. Il est donc proposé de mettre en place une taxe sur les appareils les plus haut de gamme, dont la hausse continue du prix n'effraie pas les consommateurs concernés.

Nous prônons une baisse de la pression fiscale en France et non la création de nouvelles taxes. Encore une fois, le tempo ne me paraît pas particulièrement approprié. En revanche, une réflexion au titre des investissements d'avenir et de ce que veut la France en matière d'ambition numérique serait opportune. La commission émet donc un avis défavorable

permettant de favoriser le développement du marché mahorais, notamment caractérisé par le plus faible taux de couverture de France, très significativement inférieur aux autres territoires, et le plus faible niveau de vie de France. Le

Bien que présentés comme « inefficients » par ce projet de loi de finances, ces mécanismes de réduction de l'impôt sur le revenu et sur les sociétés sont au contraire complémentaires du crédit d'impôt dont bénéficient les organismes de logements sociaux.

dotés aux réserves impartageables pour la réserver aux versements aux réserves impartageables dépassant les dotations obligatoires en application des articles 16 et 19 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. La loi impose aux SCIC de verser 15 % de leurs résultats en réserve légale et au minimum 50 % des résultats, dans des réserves impartageables, après déduction du versement à la réserve légale. En pratique, les SCIC versent la quasi-totalité de leurs résultats en réserves, car il s'agit pour elles de constituer ainsi des quasi-fonds propres indispensables à leur croissance. L'administration a dû estimer que ce dispositif était sous-utilisé, concernant plus de 800 sociétés pour un coût fiscal d'environ 1,6 million d'euros. Cependant, cette « sous-utilisation » est liée non à une inutilité, mais à la relative jeunesse du statut, créé en 2001 et consolidé par la loi relative à l'économie sociale et solidaire de 2014, avec une forte croissance- surtout depuis 2012 -et un essaimage dans de nombreux secteurs d'activités. Le Gouvernement soutient d'ailleurs leur expansion comme mode d'entreprendre conciliant activité économique et intérêt général, notamment dans les domaines de la lutte contre les déserts médicaux- sujet très important actuellement -, le développement de l'énergie citoyenne et de l'habitat partagé- notamment les coopératives HLM -, la mutation du secteur du sport ou la revitalisation des territoires. Les collectivités elles-mêmes s'impliquent très fortement dans le développement des SCIC, reconnaissant leur fort impact territorial. À ce titre, 40 % des SCIC ont une ont une ou plusieurs collectivités locales, principalement du bloc communal, à leur capital. Elles créent des activités et des emplois sur les territoires, tout en ayant la particularité d'associer les parties prenantes à la gouvernance et de réinvestir leurs excédents dans leur projet économique et social. La suppression de la déductibilité de 57,5 % des sommes mises en réserves impartageables, correspondant aux réserves obligatoires du fait de la loi, stopperait net la croissance des SCIC existantes en mutation et remettrait en cause la création de SCIC ou la transformation d'associations, alors même qu'il s'agit d'un moyen privilégié d'évolution de leur modèle économique. C'est pourquoi il est proposé de conserver le dispositif existant, qui permet aux SCIC de financer leurs investissements, et, ainsi, de réaliser leur mission d'utilité sociale et d'intérêt collectif.

et voté par de nombreux groupes à l'Assemblée nationale, vise à revenir sur une disposition du projet de loi de finances initial limitant une mesure d'aide fiscale accordée aux SCIC en matière d'impôt sur les sociétés. Toutefois,

217 du CGI, qui permet de défiscaliser les logements loués dans le respect des plafonds de loyers et de ressources prévus au dispositif du prêt locatif social. Jusqu'à présent, le bénéfice de l'article 217 était ouvert aux bailleurs privés soumis à l'impôt sur les sociétés pour leurs programmes de logements sociaux. Le Gouvernement justifie cette mesure par le fait que les organismes de logement social établis dans un département d'outre-mer bénéficient déjà d'un crédit d'impôt pour la réalisation et la réhabilitation de leur parc locatif social, l'article 244 X du CGI. Or, contrairement à l'article 217 , l'article 244 X n'ouvre droit à l'aide fiscale qu'aux organismes de logement social et non aux bailleurs privés pour leurs programmes de logements sociaux. Cet amendement vise donc à rétablir les dispositions de défiscalisation de l'article 217 à destination des bailleurs privés soumis à l'impôt sur les sociétés pour leurs programmes de logements sociaux

sur les neuf amendements identiques, qui visent à préserver la situation des SCIC. Un mot d'explication : il se trouve qu'à l'Assemblée nationale l'article 11 a été supprimé après l'adoption d'un amendement de suppression ; la seconde délibération avait pour objectif de rétablir l'article. Or ce rétablissement a

à un montage en défiscalisation, donc des contribuables qui décident de financer ce type d'opération, vous élaborez des financements de 100 000, 150 000, voire 200 000 euros,

uniquement au crédit d'impôt. En d'autres termes, le logement social privé ne pourra désormais être financé que par des bailleurs sociaux qui, s'ils ont un chiffre d'affaires de 20 millions,

Par conséquent, si, au moment de l'agrément, on arrivait à dire que ce crédit d'impôt est une créance, qui peut être nantie ou faire l'objet d'une mobilisation commerciale, oui, on pourrait le financer- non plus à taux zéro, comme le Gouvernement s'y était engagé. Aujourd'hui, vous supprimez tout

absurdes. Ce qui est absurde, c'est de faire financer le logement social des organismes d'intérêt public que sont les organismes HLM par des crédits d'impôt ou même

la seule condition posée étant que ces dépenses n'aient pas été effectivement déduites des revenus. Un tel cumul d'avantages serait extrêmement coûteux. Par

Le 6 septembre 2017, la collectivité de Saint-Martin a été frappée par l'ouragan Irma, qui a dégradé près de 95 % de ses infrastructures. Depuis Depuis maintenant plus d'un an, l'île de Saint-Martin est entrée dans une phase de reconstruction. La réussite de cette phase étant conditionnée à la redynamisation des secteurs productifs du territoire, la collectivité de Saint-Martin a plus que jamais besoin d'incitations fortes, destinées à attirer les capitaux des investisseurs français désireux de contribuer à la réactivation économique de l'île.

cinq ans, au même rang que la Guyane et Mayotte afin que les investisseurs français, au sens de l'article 199 B du code général des impôts, puissent bénéficier du taux de réduction d'impôt majoré de 45,9 % au lieu du taux de droit commun de 38,25 % applicable en matière d'investissement productif.

dans le cadre des engagements pris- et tenus ! De même, nous avons versé par anticipation un peu plus de 10 millions d'euros de dotations. L'État répond donc présent pour la reconstruction. Il ne considère pas qu'il soit opportun de jouer sur des mécanismes de défiscalisation.

Le langage utilisé pour la communication est parfois particulièrement gênant. J'ai ainsi entendu dire, lors du dernier voyage du Président de la République dans nos îles,

aujourd'hui, le port du Marin est devenu la référence de la Caraïbe en matière de plaisance et de nautisme. Je dis bien : la référence ! Des bateaux se détournent de partout dans la Caraïbe pour venir

Mes chers collègues,

le gouvernement du Royaume des Pays-Bas vient d'injecter une somme importante pour la réhabilitation et la reconstruction de Sint Maarten. Imaginez ce que ressentent les citoyens français de l'autre côté de la